La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 10 juin 2020 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. M. Martial Bourquin a fait connaître à la présidence qu'il se démettait de son mandat de sénateur du Doubs à compter du lundi 15 juin 2020, à minuit. En application de l'article L.O. 320 du code électoral, il est remplacé par Mme Marie-Noëlle Schoeller, dont le mandat de sénatrice a commencé aujourd'hui, à zéro heure. En votre nom à tous, je souhaite la plus cordiale bienvenue à notre collègue. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires est parvenue à l'adoption d'un texte commun. Mes chers collègues, par lettre en date du 15 juin, le Gouvernement demande de compléter l'ordre du jour du mercredi 17 juin par la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. En conséquence, nous ne siégerons pas jeudi 18 juin.

Mme la ministre des outre-mer. Madame la ministre, ma question porte sur le traitement des listes électorales par l'État en Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est engagée depuis vingt-deux ans dans le processus de l'accord de Nouméa, qui se conclut par trois référendums d'autodétermination, dont le premier a eu lieu le 4 novembre 2019 et a donné une majorité claire pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. Lors de ce premier scrutin, les personnes de statut coutumier et les personnes de droit commun nées en Nouvelle-Calédonie avaient été traitées de la même manière, à savoir qu'elles avaient été inscrites de manière automatique sur les listes électorales. Cependant, pour le deuxième scrutin, cette disposition n'est plus valable et seules les personnes de statut coutumier, c'est-à-dire les Kanaks, pourront être inscrites automatiquement, les natifs de droit commun devant effectuer des démarches complexes et fastidieuses pour s'inscrire. Lors du comité des signataires du 10 octobre 2019, devant l'opposition de l'ensemble des partis loyalistes, le Gouvernement s'est engagé à faire le nécessaire pour que 100 % des natifs soient inscrits afin qu'il n'y ait pas de différence avec les inscriptions automatiques de Kanaks. limite d'inscription du 31 décembre 2019, l'objectif des 100 % était loin d'être atteint. Cette situation était dénoncée publiquement par les présidents de groupe majoritaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, par la présidente de l'Assemblée de la province Sud et par le président du gouvernement local. j'aimerais connaître les mesures envisagées pour lutter contre cette discrimination, qui ouvre à un risque de résultat favorable à l'indépendance en raison d'un traitement inéquitable des listes électorales par l'État et à une contestation du résultat.

Comme vous l'avez rappelé également, il existe une liste électorale spéciale pour ce référendum. Il a été décidé, lors des comités des signataires du 5 juin 2015 et du 2 novembre 2017, de dispenser certaines catégories d'électeurs de toute démarche pour être inscrits sur la liste « spéciale consultation ». En effet, cette faculté n'a pas été étendue au deuxième référendum. C'est sur proposition du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et à la quasi-unanimité- 52 voix sur 54 -, qu'a été adoptée la proposition de réserver ce cas très particulier à la seule première consultation. C'est donc bien pour tenir compte du consensus exprimé localement par cette assemblée que nous avons modifié notre projet initial.

il ne s'agit pas de personnes, car l'absence de numéro unique d'identification en Nouvelle-Calédonie rend effectivement délicate l'identification des personnes physiques. Au final, sur 1 053 identités absentes des listes électorales, mais se retrouvant sur des fichiers sociaux- les données

Classée en zone de sécurité prioritaire, la commune souffre d'une baisse constante des effectifs de ce poste de police depuis plusieurs années, conduisant inéluctablement à la présence insuffisante d'agents sur le terrain. cette insuffisance d'effectifs pour lutter contre un sentiment d'insécurité accru depuis le meurtre d'un jeune homme de 18 ans, en mai 2019, un événement dramatique et violent qui a marqué tout le monde. Le maire, en outre, m'a fait part de nombreuses autres difficultés. Les prises de poste par les agents de police d'Hérouville-Saint-Clair à Caen, la commune voisine, tous les matins et tous les soirs, diminuent d'une heure au moins la présence sur place des policiers. Du coup, les heures d'ouverture et de fermeture du poste ne répondent pas aux besoins d'une ville comme la sienne, qui, je le rappelle, est classée en zone de sécurité prioritaire. Par ailleurs, les agents de police nationale se voient assigner des missions supplémentaires qui ne relèvent pas de leurs attributions, comme le transfert vers le centre de rétention administrative de Rouen. Enfin, les mises à disposition des personnes auteures d'infractions au commissariat de Caen par les agents de la police municipale, plutôt qu'à celui d'Hérouville-Saint-Clair, en vertu de l'article 73 du code de procédure pénale, constituent un véritable problème. En effet, cette situation nuit à la nécessaire proximité de l'action publique en matière de sécurité on agit et on prend en charge sur place. Là, le message est évidemment beaucoup plus clair. Tous ces éléments avaient été indiqués lors du dépôt de cette question en novembre 2019. Or j'ai eu la confirmation, il y a encore quarante-huit heures, que, depuis lors, rien n'avait changé.

Madame la sénatrice de la Provôté, en l'absence de mon collègue Laurent Nunez, je vais vous lire sa réponse. Nous partageons les mêmes objectifs, madame la sénatrice : renforcer la présence des policiers sur le terrain et lutter sans relâche contre la délinquance. Cela correspond à la fois aux attentes légitimes de nos concitoyens et, bien sûr, à la politique mise en oeuvre par le ministère de l'intérieur depuis près de vingt mois maintenant. Pour preuve que les policiers sont bel et bien mobilisés au contact de la population, je souhaite vous donner un seul chiffre 11 000 heures ont été consacrées à des missions de voie publique par les policiers d'Hérouville-Saint-Clair en 2019. Par ailleurs, le Gouvernement se félicite aussi du travail mené avec la police municipale : la signature, en décembre 2019, d'une nouvelle convention de coordination entre cette dernière et la police nationale témoigne d'un partenariat vivant et dynamique, et s'inscrit dans notre volonté visant à favoriser un continuum de sécurité. S'agissant de votre question relative aux effectifs du commissariat, je tiens d'abord à souligner que la circonscription de police de Caen à laquelle est rattachée Hérouville-Saint-Clair s'appuie à ce jour sur 464 agents, alors que son effectif était de 459 agents à la fin de 2016. Elle bénéficie en outre d'un nombre de gradés et de gardiens supérieur de 6 à son effectif de référence. Quant au commissariat subdivisionnaire d'Hérouville-Saint-Clair, son effectif est aujourd'hui de 24 agents, identique à ce qu'il était il y a un an.

Au-delà, la présence est assurée chaque fois que nécessaire par des unités de la circonscription. Quant à la mise à disposition des personnes interpellées par la police municipale à Caen plutôt qu'à Hérouville-Saint-Clair, elle répond à un impératif opérationnel : permettre aux fonctionnaires de se concentrer sur des missions d'enquête et de terrain plutôt que sur des missions de et de tâches purement procédurales qu'impliquerait la gestion des mises à disposition. Le nombre de personnes mises à disposition par la police municipale n'est pas assez significatif pour justifier une exception. La mobilisation de la police nationale est donc bien réelle, madame la sénatrice. Elle a porté ses fruits en 2019 : le commissariat a enregistré une baisse des principaux indicateurs de la délinquance, notamment une baisse de 11 % des violences physiques, de 40 % pour les seules violences physiques crapuleuses, et de 30 % des atteintes aux biens.

Madame la ministre, à l'heure où nos policiers et gendarmes ont besoin d'un soutien sans faille de nous tous et de la République, alors que les situations où ils sont mis en danger s'accroissent, il apparaît plus que jamais nécessaire, indispensable, j'oserais même dire vital, de mettre en oeuvre les moyens budgétaires, mais aussi organisationnels qui les protègent et renforcent leur efficacité, notamment en zone de sécurité prioritaire. Cela mérite quand même d'être regardé avec une plus grande attention. Si une zone est dite prioritaire, cela doit se traduire par les effectifs réels sur le terrain, un temps permanent de présence sur le terrain, et une et une présence qui soit à la fois dissuasive et active. Et pour assurer une présence dissuasive, il faut être sur place ! Une zone de sécurité prioritaire, c'est un contenu. À Hérouville-Saint-Clair comme ailleurs, un bilan doit être fait

Même si ce nombre est en baisse depuis dix ans, il reste néanmoins très élevé. Certes, dans beaucoup de cas, ces accidents sont essentiellement dus au comportement inapproprié des usagers. Mais il est possible de résoudre ce problème grâce à un système de détecteurs d'obstacles sur passage à niveau automatique, appelé Dopna. Il existe un process breveté par l'École centrale de Lille, dont le coût est estimé à environ 50 000 euros par installation. Celui-ci a été expérimenté par SNCF Réseau sur Lille il y a plus de deux ans et, depuis lors, nous n'avons aucune réponse, alors que l'on teste des systèmes étrangers d'un coût cinq ou six fois supérieur.

? La parole est à Mme la secrétaire d'État. Monsieur le sénateur Dany Wattebled, vous avez appelé l'attention de mon collègue Jean-Baptiste Djebbari sur la question de la sécurisation des passages à niveau du réseau ferré national. C'est un point très important, et voici les éléments que je peux partager avec vous. Vous l'avez souligné, les accidents aux passages à niveau sont la deuxième cause de mortalité sur les lignes ouvertes à la circulation des trains. Des accidents tels que celui d'Allinges en 2008, celui de Millas en décembre 2017, nous le rappellent malheureusement trop douloureusement. La sécurisation des passages à niveau est un impératif auquel le Gouvernement fait face avec détermination. C'est l'objectif même d'un plan d'action annoncé le 3 mai 2019, dont la mise en oeuvre a d'ores et déjà fait l'objet d'un premier bilan, que Jean-Baptiste Djebbari a dressé en novembre dernier. Ce plan est décliné en quatre axes et dix mesures fortes. Il vise à renforcer la connaissance des passages à niveau et du risque, qui est un préalable, à accentuer la prévention et la sanction, à amplifier la sécurisation par des mesures d'aménagement et à instaurer une gouvernance nationale et locale pour mieux piloter cette politique. Je tiens à souligner qu'en complément de ces grandes orientations, le plan s'appuie sur une augmentation de 40 % des crédits d'État d'ici SNCF Réseau expérimente, dans le cadre d'une des mesures de ce plan, un dispositif de détection de la présence d'obstacles qui traversent des voies et qui sont susceptibles de déclencher l'arrêt des circulations. Cinq passages à niveau bénéficient d'un radar de technologie Lidar. La détection d'un véhicule doit aussi activer, sans perdre une seconde, le freinage d'urgence du train qui approche. Les résultats de cette expérimentation ne sont pas encore connus, mais ils permettront de déterminer les suites à donner. Vous évoquez dans votre question la solution dite du Dopna. Loin d'être automatique, ce dispositif repose en fait sur le recours à une caméra observée par un opérateur. Il ne garantit donc pas le niveau de réaction exigé en cas de détection d'un incident. C'est pourquoi, après avoir soutenu cette innovation Dopna en 2015, SNCF Réseau a décidé de ne pas aller plus loin. Je précise aussi que le chiffre de 50 000 euros par passage à niveau qui a été cité n'inclut pas le coût du dispositif de transmission et de gestion d'alerte, ce qui ne permet pas d'établir une bonne comparaison. Pour conclure, je rappelle que la loi d'orientation des mobilités intègre plusieurs dispositions nouvelles, telles que l'obligation de réaliser un diagnostic de chaque passage à niveau, l'obligation de prévenir les usagers de la route que leur itinéraire traverse un passage à niveau.

chargé des transports. Madame la secrétaire d'État, je voudrais revenir sur le protocole d'itinéraire sur la RN 20, en Ariège. Ce protocole a été signé le 22 mars 2017 par Bernard Cazeneuve, Premier ministre, le préfet de la région Occitanie, la présidente de la région Occitanie et le président du département de l'Ariège. Il précise un projet global d'aménagement de cet itinéraire et identifie les opérations prioritaires et leur financement. Il comprend également un volet d'accord international entre la France et Andorre sur les travaux de sécurisation contre les risques naturels sur la RN 20 entre Tarascon et Andorre. Au final, 158 millions d'euros d'engagement ont été pris. J'avais interrogé Mme la ministre de la transition écologique et solidaire lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités sur les engagements financiers de l'État. Ceux de la région et du département ont déjà été clairement actés, à hauteur de 27 millions d'euros chacun, et le gouvernement andorran a fait de même à hauteur de 10,5 millions d'euros. Dans sa réponse, la ministre m'avait assuré qu'elle resterait « attentive, dans le cadre de la programmation des contrats de plan État-région, à ce que les engagements pris en 2017 dans l'accord franco-andorran soient honorés ». Le Président de la République a affirmé la même chose lors de son déplacement en Andorre en septembre dernier, précisant : « Je souhaite aussi que nous puissions continuer les investissements en termes d'infrastructures qui rendent plus simple l'accès à la France. Nous continuerons d'investir et nous inscrirons des crédits dans le prochain contrat pour continuer d'élargir la route nationale, de procéder aux travaux qui permettront de rejoindre plus rapidement Andorre et de sécuriser l'accès. Or, aujourd'hui, un flou subsiste quant à l'intégration de ces travaux dans le contrat de plan État-région (CPER) à venir, d'autant que Mme Borne précisait, lors d'une audition devant la commission des affaires économiques sur la loi de

quand la participation financière de l'État sera enfin inscrite et sous quelle forme : soit une intégration dans le CPER en cours, soit une inscription dans celui qui est à venir, c'est-à-dire celui de la période 2021-2027 ? De cette réponse dépendra, bien sûr, l'engagement des travaux. Ce serait une bonne idée pour relancer l'économie en général, les travaux

Ce protocole prévoit, comme vous l'avez dit, deux modalités de financement : d'une part, la déviation de Tarascon et ses aménagements annexes, qui seront cofinancés par l'État et les collectivités au travers des contrats de plan État-région actuels et futurs à hauteur de 136,9 millions d'euros, dont 60 % de participation de l'État ; d'autre part, les travaux de sécurisation contre les risques naturels, qui sont, eux, cofinancés à parts égales par la France et par Andorre à hauteur de 21 millions d'euros grâce à un accord international publié en juillet 2018. À ce jour, les financements disponibles sont, d'une part, 3,5 millions d'euros inscrits au CPER Occitanie 2015-2020 pour mener les études de la déviation de Tarascon et ses aménagements annexes, et, d'autre part, 5 millions d'euros correspondant aux deux premières années d'engagement de l'accord franco-andorran. En 2020, 2 millions d'euros ont été affectés afin de mener diverses études, notamment des sondages géotechniques pour le tunnel de Quié et pour acquérir le foncier nécessaire aux travaux.

de mener les premiers travaux dès 2019 avec l'installation de filets paravalanches, de filets pare-blocs, de panneaux à messages variables, la création d'une aire de chaînage et l'étude du paravalanche H2, élément important de l'accord. Ainsi, à ce jour, les engagements pris dans le cadre du protocole d'itinéraire sur la RN 20 en Ariège sont respectés. La complexité des opérations les plus importantes, comme la déviation de Tarascon ou le paravalanche H2, fait que les travaux ne pourront pas être engagés avant plusieurs années d'études. Le financement de la déviation elle-même pourra donc être envisagé dans la prochaine contractualisation « mobilité » entre l'État et les collectivités en Occitanie. En ce qui concerne le paravalanche, le financement spécifique sur le budget de l'Afitf restera disponible sur la durée pour répondre aux besoins de l'opération.

En application du règlement européen du 25 octobre 1993 relatif à l'accès au marché du transport routier, les acteurs de ce secteur, notamment l'Organisation des transporteurs (OTRE), réclament depuis deux mois l'application de la clause de sauvegarde. Le Gouvernement ne semble pas encore s'être prononcé sur cette question. Pourtant, en ce contexte de sortie de crise sanitaire, deux inquiétudes majeures sont soulevées par les professionnels du secteur. Tout d'abord, une inquiétude portant sur la santé économique des entreprises de transport routier. Alors qu'elles sont ralenties par les mesures de chômage partiel- 81 % d'entre elles sont en arrêt total ou connaissent une très forte baisse d'activité -, la reprise est lente et progressive. Il est donc crucial de leur garantir une activité minimale sans que celle-ci soit captée par des pavillons étrangers. Par ailleurs, la seconde inquiétude concerne les conditions sanitaires dans lesquelles exercent les entreprises étrangères lorsqu'elles transportent des marchandises sur le territoire national. Il apparaît que celles-ci ne seraient pas forcément aussi strictes que les mesures barrières respectées par nos conducteurs français. Ainsi, ma question est simple : quelle est la position du Gouvernement sur le sujet et celui-ci a-t-il prévu de saisir l'Union européenne afin de faire valoir la clause de sauvegarde et, donc, de suspendre le cabotage pour une période de six mois ? je vous remercie en ce qui concerne la suspension du cabotage routier, la désorganisation actuelle de l'économie a atteint la plupart des activités économiques, dont le transport routier de marchandises. Ainsi, dès le début de la crise, le Gouvernement a engagé un dialogue approfondi avec les représentants de ce secteur stratégique. Je veux réaffirmer devant vous que la nécessité d'accompagner ce secteur est totalement partagée par le ministère que je représente aujourd'hui. Le transport de marchandises a démontré son rôle majeur pour l'économie française lors de cette crise sanitaire et la reprise progressive de l'activité économique ne doit bien évidemment pas se faire au détriment de ces professionnels. Un plan ambitieux de soutien décline des dispositions pour toutes les entreprises : report de cotisations sociales et de charges fiscales, voire annulation pour les entreprises les plus fragilisées (Bpifrance) en matière de soutien à la trésorerie et de garantie de prêts bancaires ; ou encore aides directes un fonds de solidarité pour les petites entreprises. À ces mesures, qui concernent toutes les entreprises françaises, s'ajoute un soutien spécifique au secteur du transport routier

qui doit normalement être payée au plus tard le 1 septembre de cette année, est reportée de trois mois, ce qui soulagera les entreprises de 90 millions d'euros. Nous n'ignorons pas que certaines pratiques abusives, comme le cabotage systématique, contribuent à une concurrence déloyale dans un contexte déjà très difficile. Ce n'est pas tant le cabotage en lui-même qui est en cause que ses abus et- vous l'avez dit -ce sujet est d'abord européen. Le Gouvernement souhaite donc l'adoption rapide des volets « social » et « accès au marché » du paquet mobilité, car ils renforceront l'équilibre de la concurrence au sein du marché communautaire. Nous approchons du but : la commission du transport et du tourisme du Parlement européen vient d'adopter les projets de compromis qui seront examinés en séance plénière au début du mois de juillet prochain. La France aura ainsi obtenu le renforcement des capacités de contrôle et de lutte contre le cabotage systématique. Dans l'attente, le Gouvernement demeure très attentif au respect des règles en vigueur. Je tiens à rappeler que les donneurs d'ordre doivent eux aussi exercer leur devoir de vigilance en la matière. Enfin, mon collègue chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a donné instruction aux services de contrôle pour que la lutte contre les infractions au cabotage soit une priorité d'action.

Madame la secrétaire d'État, en décembre dernier, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2020, le Gouvernement a pris l'initiative de faire adopter l'augmentation de 10 millions d'euros des crédits du programme « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat ». Selon l'objet de l'amendement déposé à cette fin, le exceptionnelle et transitoire un dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018 ». On peut d'ailleurs se demander pourquoi la seule année 2018 Quelques semaines plus tard, à l'occasion de l'examen par le Sénat de ma proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, adoptée à l'unanimité le 15 janvier dernier, plusieurs sénateurs ont exprimé des interrogations sur cette initiative du Gouvernement. Celle-ci crée, de fait, un dispositif temporaire dérogatoire au droit commun et doté d'une capacité financière par ailleurs très limitée au vu de l'ampleur des sinistres engendrés par des phénomènes non reconnus de retrait-gonflement des argiles.

Pour apporter des réponses durables à ce problème majeur, qui frappe chaque année l'ensemble du territoire métropolitain, la mission a formulé plusieurs recommandations : il s'agit de faire évoluer les politiques de prévention et d'indemnisation des catastrophes naturelles.

Un amendement à la loi de finances pour 2020 a effectivement procédé à une augmentation, à hauteur de 10 millions d'euros, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement du programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat est de mettre en place, de façon exceptionnelle et transitoire, un dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018. Cette aide a vocation à être réservée aux propriétaires occupants aux revenus très modestes de bâtiments d'habitation à usage de résidence principale situés dans une commune ayant formulé, au titre de l'année 2018, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,

l'occupation. Il est en cours de calibrage. Ce travail sera fini prochainement, le plus rapidement possible, pour que les ménages puissent être indemnisés d'ici à la fin de l'année. La distribution des aides sera organisée par les préfectures des départements concernés. Il s'agit de départements dont l'intensité de la déshydratation des sols, selon les critères techniques en vigueur, n'a pas été suffisante en 2018 pour que leur territoire soit reconnu en situation de catastrophe naturelle, mais qui présentent pour autant un taux de sinistres élevé et des critères météorologiques de second rang illustrant une situation de sécheresse anormale. Néanmoins, ce dispositif reste ponctuel. Il n'a pas vocation à répondre à l'ensemble des demandes d'indemnisation. Pour progresser, le lancement d'une mission d'étude est prévu cette année ; elle aura pour objet d'apporter des solutions pérennes d'accompagnement des victimes des épisodes de sécheresse-réhydratation.

Ce projet suscite de l'inquiétude chez les habitants comme chez les élus. Ces derniers se sont regroupés en un collectif créé par Eugénie Ponthier, maire adjointe d'Épinay-sur-Seine. En janvier dernier, 104 élus de tous bords politiques ont adressé un courrier au Président de la République pour l'alerter sur les dangers de l'extension de l'aéroport. Si ADP a annoncé un report de la consultation publique à l'automne 2020, il n'a pas donné de date précise à ce jour ; or il est essentiel que cette consultation ait lieu, car les citoyens, notamment les riverains de l'aéroport, directement touchés, doivent pouvoir s'exprimer sur ce projet.

ne peut qu'accentuer. Ce type de projet a un impact considérable sur l'environnement et sur le climat. Le terminal 4 entraînerait une augmentation de 40 % du trafic aérien, soit plus de 500 vols journaliers supplémentaires, couplée à une densification prévue des terminaux existants. Le chiffrage des émissions de CO2 annoncé par ADP ne prend en compte que les phases de roulage, de décollage et d'atterrissage. Mais les avions effectuent aussi des trajets dont la France est pour partie responsable. Le Haut Conseil pour le climat préconise de les prendre en compte dans notre objectif de neutralité carbone. En incluant la moitié des trajets, 15 millions de tonnes d'équivalent CO2 s'ajouteraient aux émissions annuelles de la France d'ici à 2037. également inclure les augmentations de trafic routier pour accéder à l'aéroport par l'A1 et l'A3, déjà surchargées. Enfin, ce projet n'est évidemment pas sans lien avec la volonté de privatiser ADP et de réaliser le Charles-de-Gaulle Express pour quelque 20 000 usagers journaliers, alors que les transports du quotidien, comme le RER B, souffrent de sous-investissement. Le trafic aérien a subi un choc massif avec la pandémie de Covid-19. Nous avons là une occasion de repenser notre modèle de consommation et de production. Saisissons-la ! Madame la secrétaire d'État, l'urgence environnementale est là : allez-vous vous opposer à ce projet nocif ? La

dans la transition énergétique et écologique. C'est d'ailleurs l'esprit qui nous a animés pour la mise en oeuvre du plan de relance appliqué au secteur aéronautique. Les opérateurs du transport aérien sont déjà soumis à différents dispositifs contribuant à la lutte contre le changement climatique, dont la mise en oeuvre est une priorité du Gouvernement. Je pense par exemple à l'entrée en vigueur du dispositif dit Corsia, mécanisme mondial imposant dès 2021 la compensation de la croissance des émissions de carbone des vols internationaux. Les réflexions engagées à l'échelle européenne dans le cadre du Pacte vert visent aussi l'accélération de la transition énergétique du transport aérien, avec le développement des carburants aéronautiques durables ou le renforcement des dispositifs en place comme le marché carbone européen.

Par ailleurs, la crise sanitaire affecte les perspectives de croissance de moyen terme du trafic aérien. Les niveaux de trafic de 2019 pourraient ne pas être atteints avant 2023. Dans ce contexte, le calendrier du nouveau terminal 4 de Paris-Charles-de-Gaulle fera l'objet d'un réexamen. soyez certain que la maîtrise de tous les impacts environnementaux liés à l'activité de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle est une priorité. Le Gouvernement veillera à ce que les nuisances sonores, les émissions de polluants et leurs effets sanitaires soient maîtrisés. En particulier, l'étude dite « d'approche équilibrée », qu'Aéroports de Paris va mener en 2021, devrait permettre de progresser dans la prise en compte de la problématique du bruit, notamment la nuit.

Ils ont, de ce fait, visé l'Union européenne. En conséquence, à l'automne 2018, les négociations entre le président des États-Unis et celui de la Commission européenne ont entraîné une augmentation de 112 % de l'importation de soja américain par l'Union européenne. européenne. La Commission européenne essaie de limiter la production européenne de biocarburants de première génération, et il semblerait que l'importation de soja ait été permise à cette même fin. Cette décision commerciale apparaît comme un coup porté à la production de matières premières pour les biocarburants au sein de l'Union européenne, et les agriculteurs français ne comprennent pas cette mesure. Quant à l'Union européenne, elle ne peut choisir de remplacer l'huile de palme par une matière première tout aussi nuisible à l'environnement. On sait que le soja est également utilisé pour nourrir les bêtes destinées à produire de la viande. À ce sujet, Emmanuel Macron a indiqué en 2019 vouloir une souveraineté protéinique de la France. Ainsi, comment expliquer la position européenne, qui va à l'encontre de la déclaration du Président de la République et des objectifs européens en matière d'environnement, d'énergie et d'agriculture ? Pourriez-vous nous indiquer la position française sur ce sujet ? La

développement durable en prend un coup ... De son côté, l'Union européenne prend ses décisions comme elle l'entend. Elle fixe un cadre très clair pour les biocarburants. Ainsi, pour contribuer aux objectifs d'énergies renouvelables, les biocarburants doivent respecter les critères de durabilité fixés par la directive sur les énergies renouvelables de 2009. Ces critères portent tant sur la production de biomasse que sur les gaz à effet de serre dégagés sur toute la chaîne de production. Ils seront d'ailleurs renforcés en 2021. C'est la raison pour laquelle la France s'inscrit dans le cadre des décisions de l'Union européenne. Le 29 janvier 2019, la Commission européenne a reconnu le système de certification de la production du soja américain comme étant compatible avec les normes de durabilité de l'Union européenne. La reconnaissance de ce système facilite l'incorporation de soja américain dans les carburants européens. Cela n'était nullement interdit auparavant. Mais c'est parce que nous considérons que les biocarburants issus de soja certifié durable peuvent contribuer aux objectifs d'énergies renouvelables dans les transports qu'une telle

de l'article 24 de la loi Éthique et transparence du sport professionnel du 1 mars 2017. Toutefois, ce dispositif se révèle insuffisant : il est désormais nécessaire de renforcer les mesures protégeant les ayants droit et diffuseurs et d'assurer une lutte enfin effective contre le piratage des contenus sportifs en direct. La valeur des droits sportifs en France dépassera les 1,5 milliard d'euros dès la saison sportive 2020-2021, et ces droits sont un des éléments importants de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Le phénomène du piratage des contenus sportifs, quant à lui, connaît un véritable essor depuis plusieurs années ; le manque à gagner estimé serait de l'ordre de 500 millions d'euros et de plusieurs centaines de milliers d'abonnés. En examinant le projet de loi de réforme de l'audiovisuel, les députés ont adopté très largement en commission des affaires culturelles un article 23 visant la mise en oeuvre d'un dispositif spécifique de lutte contre le piratage du sport. L'adoption de ce dispositif équilibré a été saluée par l'ensemble des acteurs. Alors que la crise sanitaire inflige de très fortes difficultés économiques aux acteurs du sport, la mise en oeuvre rapide d'un tel dispositif serait une réponse forte au soutien des acteurs économiques concernés. Elle permettrait également de préserver les mécanismes de solidarité au bénéfice du sport amateur. Monsieur le ministre, quel est désormais votre calendrier pour l'examen de ce projet de loi, de loi, qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la session extraordinaire ? Sous quelle forme les dispositifs seront-ils adoptés ? Nous entendons parler de textes moins ambitieux que prévu, voire d'ordonnances.

Emblèmes du Paris historique, ils participent au charme des bords de Seine : ils constituent une animation touristique, une attraction culturelle, un patrimoine littéraire et historique unique qu'il faut bien sûr préserver.

ces 227 petites librairies à ciel ouvert ont fait leur entrée en février 2019 au patrimoine culturel immatériel français : c'est un premier pas vers le classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Déjà pénalisée par les gilets jaunes, puis par les grèves des transports, la profession a une nouvelle fois été durement touchée par la crise sanitaire. Il serait malheureux que ces libraires de la Seine disparaissent, alors que bien des villes dans le monde,

Mon collègue François-Noël Buffet et moi-même avons constaté, au fil des auditions et des déplacements inhérents à notre mission de suivi des lieux de privation de liberté, que l'épreuve du confinement a révélé des failles au sein de certaines prisons. Au centre pénitentiaire de Gradignan, en Gironde, les projections de téléphones, d'armes blanches ou de boulettes de stupéfiants dans les cours intérieures de l'établissement par des individus de l'extérieur ont connu une activité intense pendant le confinement, comme à l'accoutumée malheureusement. Aux alentours de la prison, ces canaux d'alimentation représentent un véritable trouble à l'ordre public et à la sécurité des riverains. À l'intérieur, ces trafics suscitent des comportements qui mettent en danger tant le personnel pénitentiaire

une équipe pénitentiaire spécialisée, avec port d'arme, autorisée à intervenir aux abords de la prison et une volonté affirmée de la part de la direction. Justement, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet la mise en place de ces équipes de sécurité aux abords immédiats des établissements. Ainsi, le centre pénitentiaire de Fresnes a entrepris la formation de ses agents avant le confinement sanitaire et la reprend avec le déconfinement. Mais, quant à elle, la prison de Gradignan n'envisage aucune création d'unité dédiée pour la surveillance des abords de ses murs avant 2022,

Pouvez-vous venir constater par vous-même la prégnance de ces trafics dans la prison de Gradignan et entendre les représentants du personnel et le maire de la ville afin de prendre les mesures qui s'imposent ? L'attente est forte ! La parole

permet, comme vous l'avez souligné, de lutter activement contre le trafic de substances ou d'objets illicites et interdits en détention. Ces structures sécurisent les fouilles sectorielles

D'autre part, ce centre pénitentiaire va être entièrement reconstruit, avec une sécurisation totalement repensée, pour un investissement de près de 137 millions d'euros. Les travaux de démolition préalable ont démarré en juin dernier. Cette opération permettra de livrer un nouvel établissement de 600 places, entièrement sécurisé

de la justice. Monsieur le sénateur Sueur, la restitution des avoirs criminels confisqués dans le cadre des procédures pénales dites des biens mal acquis est effectivement un enjeu majeur ; elle participe à l'oeuvre de justice en faveur des populations lésées. En l'état de notre droit, les règles de restitution ou de partage ne prévoient pas un retour systématique et intégral de ces biens aux États et populations lésés. En effet, aucun mécanisme de contrôle ne garantit le bon emploi des fonds restitués, notamment leur redistribution aux populations civiles.

pays concerné. Vous n'ignorez pas les enjeux budgétaires et diplomatiques qui doivent être pris en compte. Du point de vue judiciaire, nous devons également veiller à bien délimiter le champ des infractions et à articuler le futur dispositif avec les règles habituelles d'indemnisation des victimes.

que le Premier ministre a annoncé, en juillet 2018, la fusion de Cap emploi et Pôle emploi en un lieu unique de droit commun pour les personnes en recherche d'emploi, des temps de concertation et de travail ont été organisés pour réfléchir aux modalités de rapprochement des deux entités. dans le cadre de ces réflexions consiste en un rapprochement opérationnel, Cap emploi devenant un service au sein de Pôle emploi, chargé spécifiquement de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, que le handicap soit installé, consécutif à un accident de la vie ou médical. Cette réorganisation se met en place avec des unités pilotes dans chaque région ; des expérimentations sont menées pour évaluer le nouveau dispositif en amont de sa généralisation. en amont de sa généralisation. Le maintien dans l'emploi, aujourd'hui de la compétence de Cap emploi mais pas de Pôle emploi, est un volet important et indispensable de l'accompagnement dans l'emploi des salariés en situation de handicap.

En ce qui concerne le rapprochement des deux opérateurs Cap emploi et Pôle emploi, le Premier ministre a appelé de ses voeux un lieu unique d'accompagnement aux fins, justement, de servir encore mieux les personnes en situation de handicap et de les rapprocher des entreprises.

Avec la crise économique, les entreprises sont parfois frileuses à embaucher pour la rentrée de septembre. Combien de promesses de stage, d'embauche en CDI, en CDD ou en apprentissage ont-elles été remises en question ? Combien de postes n'ont-ils pas été ouverts à la suite du confinement ? Une génération entière est en train d'être abandonnée au bord de la route ! De fait, des milliers de jeunes sont bloqués, dans l'attente de démarrer enfin leur vie professionnelle.

très petites, petites et moyennes entreprises, qui sont les premiers employeurs d'apprentis. Pourtant, l'apprentissage, nous le savons, est une chance incroyable pour les jeunes : il permet à nombre d'entre eux d'acquérir une qualification et des compétences qu'ils ne pourraient pas obtenir dans un autre cadre. Madame la ministre, depuis l'inscription à l'ordre du jour de ma question, un dispositif de 5 000 euros pour les mineurs et de 8 000 euros pour les majeurs a été adopté ; je le salue, mais je pense qu'il faut aller plus loin encore, en diminuant le reste à charge pour les entreprises

rattraper » ceux qui ont été en difficulté. Plus que jamais, nous pensons que l'apprentissage est une voie d'excellence, une voie de réussite ; plus que jamais, l'emploi des jeunes est pour nous une haute priorité. Nous aurons l'occasion d'y revenir à l'issue de la concertation en cours, mais ne doutez pas que, pour moi, c'est la première priorité de notre plan de relance de l'emploi

notamment en Seine-Saint-Denis, pour trouver un contrat en alternance au sein d'une entreprise. De nombreux jeunes, en particulier après le bac, sont contraints de renoncer à leur projet d'étude en alternance dans le supérieur, faute de trouver une entreprise pour les former et les rémunérer à temps partiel dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Trouver un contrat en alternance est un véritable parcours du combattant pour ces jeunes, dont les parents ne disposent pas toujours du capital culturel et économique nécessaire pour les aider dans leur recherche. Sans compter que les organismes de formation ne leur apportent aucun soutien, bien que certains vantent dans leur plaquette promotionnelle l'aide à la recherche que permettrait leur gigantesque réseau-

de 25 000 à 40 000 euros hors taxes, à compter du 1 janvier 2020. Or la crise sanitaire qui a secoué le pays a gravement fragilisé le tissu économique français, imposant à tous les acteurs, économiques et politiques, d'user de ressources pour s'adapter à cette situation inédite.

permettrait notamment de passer plus facilement des contrats relatifs aux travaux de voirie ou de rénovation et de favoriser, peut-être, des entreprises locales, non par clientélisme mais par souci de préserver des emplois sur nos territoires. La parole

le soutien aux acheteurs et aux opérateurs économiques confrontés aux difficultés découlant de l'état d'urgence sanitaire est l'une des priorités du Gouvernement. L'ampleur inédite de cette crise nous a d'ores et déjà conduits à adapter temporairement les règles de la commande publique, levier important de croissance et de relance de l'activité économique, tant pour la trésorerie des entreprises que pour le fonctionnement de nos services publics. Ainsi, nous avons adapté les modalités de conclusion des contrats publics pour garantir la satisfaction des besoins des autorités contractantes pendant la crise sanitaire. Afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement pour les autorités, nous avons autorisé celles-ci à prolonger les contrats arrivant à échéance pendant l'état d'urgence sanitaire. Sauf urgence, les délais de réception des candidatures et des offres ont été prolongés : les autorités ont ainsi pu aménager autant que nécessaire les modalités de participation aux procédures en cours. nous avons protégé les entreprises titulaires de contrats publics mais qui n'étaient pas en mesure de les exécuter. Lorsque l'exécution du contrat est impossible, son titulaire ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer des pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif. nous avons aidé les entreprises dont le contrat public était affecté par l'état de crise sanitaire. Afin de limiter les besoins de trésorerie des entreprises, nous avons permis aux titulaires de marchés d'aller au-delà de ce que la loi permet actuellement en termes d'avances. Par exemple, les avances financières versées aux titulaires de marchés peuvent être portées au-delà de 60 % du montant total. Toutefois, l'impératif de sécurité juridique qui nous guide et qui conditionne la réussite de la relance de notre économie impose de concilier les mesures de simplification avec nos principes constitutionnels d'accès à la commande publique.

qui font la richesse de tous nos territoires. Ils garantissent la vitalité de nos départements, mais ils sont aussi des acteurs essentiels de la formation et de l'apprentissage auxquels faisait référence à l'instant Mme la ministre du travail, Muriel Pénicaud.

En effet, les problèmes liés à l'accroissement du démarchage téléphonique sont majeurs et vont parfois bien au-delà de la simple protection du consommateur. Nous savons que nombre de nos concitoyens renoncent à répondre au téléphone, épuisés par ces appels à répétition. La nécessité de lutter contre ces appels intempestifs n'est pas nouvelle. Le dispositif Bloctel permet en théorie au consommateur de s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au au démarchage téléphonique. Or nous constatons que ce dispositif est malheureusement très inefficace. C'est pourquoi je me félicite de cette proposition de loi votée et améliorée par le Sénat, notamment par l'instauration d'un identifiant d'appel obligatoire sous forme de préfixe, qui permettra de repérer l'appel comme étant un démarchage. Je regrette cependant qu'une proposition majeure de mon groupe n'ait pu être adoptée. Elle prévoyait que, « pour que quelqu'un soit démarché par téléphone, il faut qu'il ait formulé son consentement de façon claire et explicite pays d'Europe, dont l'Allemagne, l'Autriche ou encore le Portugal, ont adopté une telle disposition, qui s'applique déjà pour les courriels et les SMS- elle est d'ailleurs tout à fait conforme au règlement général sur la protection des données.

d'un démarchage téléphonique intempestif et intrusif, l'article L. 223-1 du code de la consommation interdit à un professionnel, sous peine d'une amende de 75 000 euros, de démarcher par téléphone des consommateurs inscrits sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Ce dispositif compte aujourd'hui 4 millions d'inscrits. En moyenne, chacun des près de 10 millions de numéros inscrits sur cette liste d'opposition au démarchage est retiré chaque semaine de six listes de téléprospection, soit autant d'appels évités. Pour autant, les nuisances perdurent pour nombre de nos concitoyens, signe que de trop nombreuses entreprises ne respectent pas la loi. Le Gouvernement a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage téléphonique abusif. Ainsi, il a demandé au Conseil national de la consommation d'établir un état des lieux des pratiques de démarchage téléphonique et de proposer des mesures pour mieux lutter contre les appels téléphoniques non sollicités et la fraude aux numéros surtaxés. Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif, une proposition de loi, que vous avez évoquée, monsieur le sénateur Yannick Vaugrenard, vise à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux. Après avoir été examinée par l'Assemblée nationale, elle vient d'être adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 4 juin dernier. Prochainement, une commission mixte paritaire sera chargée de se prononcer sur les dispositions restant en discussion. Comme l'a indiqué ma collègue Agnès Pannier-Runacher, qui suit attentivement ce dossier, une fois adopté, ce texte rendra plus dissuasives les sanctions encourues en cas de non-respect du dispositif d'opposition au démarchage téléphonique et améliorera l'information des consommateurs sur leur droit de s'opposer à ce mode de sollicitation commerciale. S'il est adopté sur ce point, il devrait également introduire une interdiction du démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique. Par ailleurs, comme vous le savez, le ministère de l'économie et des finances, en particulier la DGCCRF, est mobilisé pour lutter contre les pratiques illégales de démarchage téléphonique. En 2019, plus de 1 000 établissements ont été contrôlés, conduisant à la sanction de 77 démarcheurs ne respectant pas le dispositif Bloctel pour un montant total d'amendes de 2,5 millions d'euros- ce montant a été triplé par rapport à 2018. En 2020, dix sanctions représentant plus de 200 000 euros d'amendes ont d'ores et déjà été prononcées.

ont vu leur activité complètement arrêtée en raison du Covid-19 et des mesures sanitaires qu'il a entraînées. Cette profession représente quelque 320 000 emplois directs et indirects dans le pays. Elle est la plus ancienne parmi les opérateurs de loisirs, distrayant chaque année toutes les régions de l'Hexagone, des plus rurales au plus urbaines. Leur présence favorise l'économie locale, en particulier la restauration. La situation des forains est d'autant plus dramatique qu'ils ont profité de la basse saison pour réviser et entretenir leur matériel. Cela représente d'importants investissements, pour certains à peine rentabilisés ou remboursés par l'exploitation de leurs installations. La désespérance a commencé à s'installer pour toute cette profession, qui a dû ranger ses manèges, alors que le calendrier des foires et des fêtes s'anime en cette période et que l'on peut légitimement s'interroger sur la possibilité de tenir la saison estivale. L'aide de l'État de 1 500 euros pour les artisans et indépendants est bienvenue.

Comme tous les professionnels, les commerçants itinérants peuvent bénéficier des mesures de soutien mises en place depuis le début de la crise. Comme vous l'avez rappelé, ils peuvent bénéficier du fonds de solidarité à hauteur de 1 500 euros, mais il ne s'agit que du premier volet. Un second volet, instruit par les régions, permet d'octroyer une aide supplémentaire. itinérants peuvent également bénéficier des mesures de soutien d'urgence mises en place pour toutes les entreprises : reports, voire exonérations de charges présentées dans le PLFR 3, prêts garantis par l'État, activité partielle pour les salariés. En outre, des aides sont proposées par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les artisans et commerçants ainsi que leur conjoint collaborateur relevant du régime complémentaire des indépendants, le

Monsieur le secrétaire d'État, je souhaite appeler votre attention sur la situation des très petites entreprises. Le 4 mai 2020, le Gouvernement annonçait une annulation des charges sociales des entreprises de moins de dix salariés qui ont été contraintes de fermer pendant la période de confinement. Je salue cette mesure, qui est une véritable aide pour ces entreprises très fragilisées par la crise. par la crise. Ce premier geste du Gouvernement est vital pour ces entreprises. Reste cependant à définir le périmètre des charges incluses, qui doit être important pour être efficace. Pour retrouver le niveau d'activité économique d'avant la crise du Covid-19, il faudra du temps. La situation sanitaire, même si elle s'améliore, reste préoccupante, et les perspectives de reprise effective sont toujours incertaines. D'après les professionnels du secteur, 400 000 très petites entreprises pourraient fermer définitivement dans les prochaines semaines. Dès lors, les dispositifs d'aide qui ont été mis en place devront durer le plus longtemps possible.

Par ailleurs, si les entreprises ayant fait l'objet de mesures de fermeture sont certes parmi les plus durement touchées, c'est toute l'économie française qui est profondément affectée. Le Gouvernement envisage-t-il d'étendre l'annulation des charges aux TPE n'ayant pas fait l'objet d'une obligation de fermeture administrative, mais qui ont vu leur chiffre d'affaires significativement diminué

qui ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pendant la période de confinement. Ce dispositif d'ampleur, qui fait partie des mesures du troisième PLFR présenté la semaine dernière, va au-delà d'une seule exonération des cotisations patronales, puisqu'une aide au paiement sera mise en place pour couvrir les autres cotisations et contributions que l'employeur doit verser. L'autre objectif de cette mesure d'exonération est de permettre une reprise rapide de l'activité des entreprises concernées en diminuant de manière massive les passifs sociaux qui ont pu être constitués durant la crise sanitaire. En effet, les TPE des secteurs ayant fait l'objet de mesures de fermeture sont celles qui ont le plus fait appel aux possibilités de report des échéances sociales depuis la mi-mars. Au demeurant, les entreprises qui auraient continué à s'acquitter de leurs cotisations et contributions sociales malgré les difficultés bénéficieront également du dispositif, ce qui constituera pour elles une aide supplémentaire pendant la période de reprise. Dans les secteurs les plus touchés, le dispositif est le plus favorable, puisqu'il portera sur un mois supplémentaire de cotisations et contributions sociales pour tenir compte du fait que les mesures de fermeture se sont souvent prolongées au-delà du 11 mai pour ces secteurs et que l'activité y sera en tout état de cause plus lente à reprendre. Par ailleurs, pour ces secteurs, le dispositif sera accessible à toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Au-delà de cette mesure, nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir les entreprises durant la phase de reprise, comme nous l'avons été durant la phase de confinement, afin de limiter les pertes d'emplois et les faillites. Si la crise affecte de façon très aiguë certains secteurs, l'ensemble de notre économie est concerné par la baisse de l'activité. C'est pourquoi le Gouvernement, tout en faisant le choix de cibler certaines de ces aides afin de garantir leur pleine efficacité au service de la reprise, met également en place des mesures de soutien à caractère plus général. Le PLFR prévoit ainsi la mise en place automatique de plans d'apurement pour les créances sociales, ainsi que la possibilité de remise de certaines dettes pour les entreprises dont l'activité aurait très fortement baissé.

remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État. Les TPE représentent deux tiers des entreprises françaises. Elles contribuent de manière non négligeable au PIB et à l'emploi sur nos territoires.

Un mécanisme de compensation a été mis en place pour les communes, mais ce dernier omettrait certaines cotisations fiscalisées par les communes, comme la contribution aux syndicats intercommunaux sans fiscalité propre,

C'est un premier couac, et je crains que ce ne soit malheureusement pas le seul dans la compensation, promise à l'euro près, de la suppression de la taxe d'habitation. Je crois qu'il est développement sur les difficultés financières des communes, qui ont été amplifiées par la crise sanitaire. En effet, la plupart des maires et des membres des équipes municipales ont dû prendre des mesures nouvelles face à cette crise, parfois en prenant le relais de l'État,

l'état actuel des choses, la compensation de leur contribution fiscalisée la taxe d'habitation au syndicat intercommunal à vocation scolaire. Ma question est donc simple : le Gouvernement compte-t-il revoir les coefficients correcteurs de transfert afin de compenser à l'euro près les pertes pour les communes de la réforme de la taxe d'habitation ? Va-t-il réparer l'oubli de la part de la cotisation syndicale

Les syndicats, qu'ils soient mixtes ou intercommunaux, sont des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre. Dès lors, ils ne disposent d'aucun pouvoir fiscal. Ils perçoivent en principe des contributions budgétaires de leurs communes membres. En vertu des alinéas 1 et 2 de l'article 1609 du code général des impôts, le comité d'un syndicat peut décider de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales, en remplacement de tout ou partie de la contribution des communes associées. Dans ce cas, les taux de fiscalité applicables à leur profit sont déterminés proportionnellement aux recettes que chacune des impositions directes locales procure à la commune. La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales augmentera mécaniquement la part des autres taxes dans le produit global communal. Toutes choses égales par ailleurs, elle se traduirait donc, du fait du mode de calcul des taux d'imposition syndicaux, par un report sur les autres impositions maintenues. Cependant, la fiscalisation des contributions communales ne peut être mise en oeuvre que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part, ainsi que le précise l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales. En d'autres termes, la fiscalisation des contributions syndicales relève d'un choix de gestion de la commune. Le syndicat étant assuré de percevoir le produit de la contribution qu'il détermine quelles que soient les modalités de financement de la quote-part attendue des collectivités membres, il n'y a pas matière à compensation pour perte de produit syndical du fait de la réforme de la fiscalité locale. La parole

avoir ce choix. Si ces compensations ne sont pas effectives, les communes vont devoir taxer d'autres acteurs- je pense particulièrement aux entreprises.

M. le ministre de l'économie et des finances. Après la crise sanitaire, notre pays est frappé par une crise économique sans précédent qui touche l'ensemble de notre économie. Secteur ô combien impacté, l'automobile a fait l'objet d'un plan de relance présenté récemment par l'État. Las, force est de constater que ce plan de soutien de l'État apporte très peu de solutions à un pan important de la filière automobile, celui de l'industrie du décolletage. Regroupant 600 entreprises et 14 000 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros, l'industrie du décolletage est confrontée à des défis majeurs. Le plan présenté ne traite que partiellement les questions de fond soulevées depuis plusieurs mois par les professionnels du secteur, et les réponses y sont inadaptées. Ainsi, qu'en est-il des contours du fonds de soutien aux entreprises, qui ne sont toujours pas clairs pour les principaux intéressés deux mois après avoir été mis en place ? Qu'en est-il du dispositif de soutien à l'emploi en discussion avec l'Union des industries et métiers de la métallurgie ? Ce plan de soutien ne suffira pas à lui seul à aider l'industrie du décolletage, déjà fragilisée par une crise structurelle avec la baisse annoncée des moteurs thermiques, l'émergence des voitures autonomes et la montée en puissance des voitures électriques. Il ne répond pas aux grands enjeux de cette industrie. Pis, il accélère une mutation des motorisations thermiques vers l'électrique, qui nécessite un volume dix fois moindre de pièces à décolleter. Les entreprises du décolletage ont toujours su prendre leur part au progrès et à l'innovation, encore faut-il que l'État les aide à passer ce cap difficile et à réussir leur mutation structurelle, comme il l'a fait pour l'automobile et l'aéronautique. L'industrie L'industrie du décolletage mérite un plan de soutien spécifique. Sans ce plan, chaque mois perdu à discuter représente environ 500 collaborateurs supplémentaires mis au chômage. Il y a véritablement urgence à maintenir ces compétences et ces emplois.

principalement des PME et des TPE familiales, qui, pour une large part, sont spécialisées dans le domaine du décolletage ou de la mécanique de précision. Les difficultés de la vallée de l'Arve ne datent pas de la crise du Covid-19. La décroissance du marché du diesel à partir de 2015 a mis en évidence les problématiques structurelles de ce secteur sa forte dépendance aux véhicules thermiques, la vieillesse relative d'une partie du système de production ainsi qu'une recherche de diversification trop modeste. La crise du Covid-19 a impacté encore plus fortement les acteurs de la vallée de l'Arve. Les entreprises tournent au ralenti, et les incertitudes sont très grandes. La plupart de ces entreprises anticipent une probable baisse de leur chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 20 % à 40 %. Les mesures d'urgence mises en place par le Gouvernement ont été massivement mobilisées par les entreprises de la vallée de l'Arve. Une part très importante de ces entreprises ont fait appel au dispositif d'activité partielle, au report de charges sociales, fiscales et bancaires ou aux prêts garantis par l'État. Si la crise actuelle aggrave encore la situation de la vallée de l'Arve, elle ne doit pas nous faire oublier les considérations de moyen et long terme, seules susceptibles d'assurer la pérennité de ces entreprises. C'est pourquoi, dans le cadre du plan de relance du secteur automobile, le nouveau fonds de soutien à l'investissement que vous avez évoqué soutiendra les projets de diversification, de modernisation industrielle, de transformation numérique, d'amélioration de la performance environnementale des sites de production ou de consolidation qui pourraient être menés par les acteurs de la filière. Des outils inédits, massifs et simples ont été débloqués pour soutenir la filière automobile et, partant, les équipementiers. Les acteurs de la vallée de l'Arve doivent mobiliser ces financements pour mener à bien leurs projets de transformation. Les moyens existent ; nous devons désormais nous en saisir au mieux pour construire le futur de la vallée de l'Arve. C'est pourquoi, en complément du plan de relance automobile, nous poursuivons également la mise en place d'un plan d'action spécifique pour soutenir la vallée en collaboration avec l'ensemble des acteurs. Plusieurs réunions ont eu lieu la semaine dernière, notamment vendredi dernier en préfecture, pour avancer avec les acteurs de la vallée. L'objectif de ce plan est de proposer des actions concrètes à prendre rapidement et qui permettront, dès la sortie de crise, de s'attaquer aux problèmes structurels de la vallée de l'Arve. Ce plan d'action doit permettre d'apporter un soutien au repositionnement stratégique des acteurs de la vallée, tout en identifiant des perspectives de diversification à moyen terme.

Elle a été l'occasion de faire un point sur la politique publique du handicap, mais aussi de préciser les jalons à venir. Cet événement illustre le fait que le Président de la République a souhaité faire de la politique du handicap l'une des priorités de son quinquennat actuel.

Sessad, cette liste d'attente compte 376 jeunes ; il s'agit de la deuxième liste la plus importante du Grand Est après le département du Bas-Rhin. Ces listes d'attente très supérieures à la moyenne dépassent l'entendement. Je peux témoigner personnellement de cette situation, car j'ai eu l'occasion de connaître du dossier d'un petit garçon de 6 ans qui devrait intégrer un IMP (institut médico-pédagogique) dans le Haut-Rhin

Il est inconcevable qu'un enfant en situation de handicap se retrouve sans autre solution. Les lacunes dans les instituts médico-éducatifs du département du Haut-Rhin concernent également le taux d'équipement.

dans notre pays, de même que nous investissons beaucoup dans l'éducation nationale, avec le ministre Jean-Michel Blanquer, pour mieux scolariser les enfants et organiser la coopération avec le secteur médico-social. Concernant la situation spécifique du département du Haut-Rhin, le taux d'équipement y est supérieur à la moyenne régionale pour les Sessad, mais inférieur en effet pour les établissements. Dans ce contexte, l'agence régionale de santé Grand Est bénéficie de financements complémentaires. À l'échelon régional, 10 millions d'euros en 2020, puis 21 millions d'euros en 2021 seront consacrés à la mise en oeuvre de solutions nouvelles. En effet, le projet régional de santé Grand Est a fixé des objectifs ambitieux en termes de parcours de personnes, en cohérence avec le mouvement de transformation de l'offre à visée inclusive et les stratégies sectorielles, notamment en matière de troubles du neuro-développement et de l'autisme. Dans le département du Haut-Rhin, la création de places en Sessad pour la prochaine rentrée figure parmi les actions prioritaires. Cet engagement, destiné notamment à venir en appui du milieu scolaire, s'est formalisé concrètement par une convention passée entre l'ARS et l'éducation nationale en juillet 2019. L'accompagnement s'organise grâce à l'engagement permanent des établissements scolaires à s'adapter aux besoins éducatifs particuliers des élèves handicapés. Ces actions seront amplifiées à la rentrée de 2020. Avec Jean-Michel Blanquer, nous allons mobiliser le comité de pilotage de l'école inclusive à la fin de cette année pour préparer cette rentrée, dans dans le prolongement de la parole forte du Président de la République lors de la Conférence nationale du handicap. Dans le département du Haut-Rhin, une unité d'enseignement maternel pour enfants autistes d'une capacité de sept places, adossée à un Sessad, sera ainsi ouverte. Enfin, pour concrétiser le principe de l'inconditionnalité de l'accompagnement de toutes les personnes handicapées et des proches aidants, un numéro d'appel national, le 0 800 360 360, et des communautés territoriales associées sont en cours de déploiement. Ce dispositif permettra de ne laisser personne, aucune famille, sans aide et de mobiliser la capacité d'innovation des associations

Vous mettez les moyens financiers, mais, concrètement, on ne les voit pas sur le terrain. Je vous demande donc, de façon tout à fait officielle, de porter une attention toute particulière à notre département. La parole

Pour autant, les effectifs n'ont pas augmenté et sont restés identiques. En outre, il n'y a pas eu, malgré la complexité des tâches et des missions, de reconnaissance salariale. En fait, se sont ajoutés

demandent le respect des missions qui étaient exigibles d'eux, l'indemnité forfaitaire de risque qui est attribuée à un certain nombre de personnels exposés,

c'est une perspective encourageante et enthousiasmante pour eux -à la catégorie B. Enfin, ils veulent des heures supplémentaires. Madame la secrétaire d'État, que comptez-vous faire face à ces revendications ?

je vous remercie pour votre question, qui me permet de vous confirmer que le CHU de Rennes respecte les dispositions réglementaires en matière d'organisation des missions attribuées à l'équipe de sécurité. Les effectifs sont supérieurs aux exigences réglementaires et aux préconisations de la commission de sécurité. Les missions exercées par l'équipe de sécurité sont prévues prévues par les textes. Leur périmètre n'évolue pas de manière continue, dans la mesure où elles ont été redéfinies depuis le 1juin 2007. Les effectifs ont été renforcés en cohérence avec l'organisation des missions, mais sont, à l'heure actuelle,

Depuis 2018, la révision de l'organisation des cycles de travail de l'équipe de sécurité intervient dans le cadre d'un dialogue social très actif. Le projet est élaboré dans le respect du principe d'équité avec les autres professionnels du CHU, afin de mieux lisser les jours de travail et de repos sur l'ensemble de l'année. Ainsi, au total, douze réunions de travail sur les deux sites et trois instances ont été organisées, afin de formaliser le recueil des avis de l'équipe comme des représentants du personnel sur le projet. La question des déroulés de carrière et des perspectives professionnelles a été abordée avec l'équipe de sécurité dès le mois de décembre 2019, afin de définir les grades cibles identifiés pour chaque fonction.

au sein de l'équipe, en lien avec les parcours professionnels de chacun. Enfin, je me permets de rappeler l'engagement permanent du CHU en termes de promotion professionnelle. Les départs en formation continue concernent plus de 3 500 professionnels non médicaux chaque année, soit plus de 50 % des effectifs.

des solidarités et de la santé. Au vu de ce qui se passe en Chine et dans le Pacifique, la réussite du déconfinement dépendra de notre capacité à tester au plus vite une grande partie de la population. la stratégie nationale de déconfinement fixe un objectif de 700 000 tests virologiques en laboratoire chaque semaine. Ces tests visent en premier lieu des personnes symptomatiques, puis, en cas de résultat positif, les individus avec lesquels elles auraient été en contact. En parallèle de ce dispositif, qui mobilisera fortement les laboratoires, il sera crucial de dépister le maximum de patients asymptomatiques. Acteurs de santé et de proximité, les pharmaciens pourraient ainsi intervenir de façon complémentaire aux laboratoires en testant l'ensemble des individus asymptomatiques qui le souhaitent, notamment ceux ayant eu des symptômes révolus durant les dernières semaines. Les tests sérologiques, on le sait, ne mesurent pas la charge virale : un individu peut donc être contagieux, même si son test sérologique est négatif. En tant que professionnels de santé, les pharmaciens auront donc pour devoir d'indiquer aux individus dont le résultat est négatif qu'ils peuvent tout de même être porteurs du virus. Ils leur rappelleront ainsi les mesures de sécurité à respecter. L'intérêt des tests sérologiques en pharmacie, menés sur la base du volontariat, est de pouvoir dépister de potentiels porteurs de virus asymptomatiques, qui ne seront pourtant pas ciblés par les tests en laboratoire. Ces tests sérologiques en officine constitueront un outil de prévention supplémentaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Avec une présence territoriale et une force de frappe- force de frappe- puisque c'est la guerre, nous dit-on ! -permettant de réaliser au minimum 500 000 tests par semaine, les pharmacies françaises représentent un levier stratégique dans le dispositif de diagnostic. La multiplication des tests sérologiques contribuera par ailleurs aux enquêtes épidémiologiques, les officines formant un réseau de poids pour enrichir la collecte et la transmission de ces informations. Ce dispositif irait dans le sens de l'avis rendu le 18 mai 2020 par la Haute Autorité de santé, qui souligne que les tests rapides d'orientation diagnostique, les fameux TROD, sont réalisables dans davantage de lieux, en comparaison avec les tests sérologiques, les TDR, réalisés en laboratoire et, bien sûr, par les professionnels de santé que sont les pharmaciens. Madame la secrétaire d'État, j'aimerais savoir ce que vous entendez faire et

Un arrêté va être prochainement pris en ce sens. Je rappelle que, dans le rapport du 14 mai sur la place des tests sérologiques rapides dans la stratégie de prise en charge du Covid-19, la Haute Autorité de santé a émis des recommandations concernant l'utilisation de ces tests par d'autres professionnels de santé que les biologistes, selon certaines indications et sous certaines conditions, notamment pour les patients ayant des difficultés d'accès à un laboratoire de biologie médicale. Tout en recommandant que les TROD soient pratiqués par des professionnels, des personnels ayant préalablement suivi une formation à l'utilisation de ce type de test du Covid-19, la Haute Autorité de santé a inclus les pharmaciens d'officine dans la liste des professionnels de santé habilités à les réaliser. De fait, les pharmacies d'officine maillent le territoire de façon très fine et contribuent à l'accès aux soins de la population.

Un mois après le début de la phase de déconfinement, au moment où les terrasses de café et de restaurant renouent avec un esprit français si convivial, plusieurs secteurs, piliers fondamentaux de notre économie, ont l'esprit moins festif et le coeur moins léger. Je veux parler de notre souveraineté sanitaire et de la situation tristement emblématique du laboratoire pharmaceutique UPSA, implanté à Agen, au coeur du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire non loin de la Gironde, UPSA, ce sont 300 millions de boîtes de médicaments vendues chaque année dans plus de 60 pays, dont 98 % de la production est réalisée et conditionnée dans le Lot-et-Garonne. UPSA, ce sont aussi 1 400 emplois directs et 3 600 emplois indirects dans mon département. UPSA, c'est une entreprise qui, au coeur même du cyclone lié au Covid-19, a pu faire face à la demande exceptionnelle en produisant et en distribuant 1 million de boîtes de paracétamol par jour. Mais UPSA, c'est aussi la triste illustration des politiques publiques industrielles contemporaines : baisse structurelle de la production, tentation de délocalisation et concurrence étrangère déloyale. S'agissant de l'industrie pharmaceutique, chaque acteur est en droit d'attendre un pilotage stratégique et une politique avantageuse en ce qui concerne le prix des médicaments « France », afin de créer un climat de confiance. En 2005, la France était le premier producteur de médicaments en Europe. Quinze ans après, nous sommes relégués au quatrième rang. La crise du Covid-19 a mis en lumière la nécessité absolue de produire en France. Pourtant, malgré la capacité avérée de ce fleuron industriel de répondre présent en temps de crise, des mesures de régulation économique, comme la baisse des prix ou la générification, sont susceptibles de pénaliser sa production en menaçant cruellement l'avenir du site situé dans le Lot-et-Garonne. Madame la secrétaire d'État, qu'envisagez-vous pour éviter des tentations de délocalisation, tout en favorisant le tissu industriel qui garantira à la France une réelle souveraineté sanitaire ?

À ce titre, tout levier incitatif permettant de développer l'investissement dans les capacités de production de principes actifs, de matières premières et de médicaments sur le territoire de l'Union européenne est examiné. Afin d'améliorer la situation, Agnès Buzyn a présenté le 8 juillet 2019 une feuille de route pour mieux prévenir, gérer et informer les patients et les professionnels de santé. Celle-ci est construite autour de vingt-huit actions et regroupée en quatre axes promouvoir la transparence et la qualité de l'information, afin de rétablir la confiance et la fluidité entre tous les acteurs, du professionnel de santé au patient ; lutter contre la pénurie de médicaments par de nouvelles actions de prévention et de gestion au niveau de l'ensemble du circuit du médicament renforcer la coordination nationale et la coopération européenne pour mieux prévenir les pénuries de médicaments ; enfin, mettre en place une nouvelle gouvernance nationale en instaurant un comité de pilotage chargé de la stratégie de prévention et de lutte contre les pénuries de médicaments. La crise du Covid-19 a confirmé le diagnostic posé et les mesures clés identifiées dans cette feuille de route. La France et, plus globalement, l'Union européenne ont vécu de manière forte la perte d'indépendance stratégique résultant de la délocalisation de la production pharmaceutique et des matières premières. La France doit rétablir ses capacités en matière de production industrielle, comme l'a rappelé le Président de la République. Produire plus, produire mieux, produire différemment sont des impératifs absolus. La France demeure très attachée à la continuité de la production de médicaments thérapeutiques aussi indispensables que le paracétamol, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19. Toutes les modalités en faveur de l'indépendance sanitaire française, de la production de la matière première aux produits finis, sont à l'étude pour garantir la continuité des traitements indispensables à l'ensemble des Français. Enfin, notre pays promeut et soutient la relocalisation, l'harmonisation et le renforcement de la coopération entre États membres pour retrouver la souveraineté européenne. Il souhaite donner un nouvel élan au travers de la mise en place d'une stratégie industrielle pharmaceutique européenne.

Néanmoins, des études ont montré que le coût d'exploitation du linge des blanchisseries hospitalières serait de 25 % au moins supérieur à celui des blanchisseries privées. En outre, l'Union des responsables de blanchisserie hospitalière (URBH) précise que 80 % d'entre elles seraient en deçà du seuil de rentabilité.

la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les bonnes conditions de travail des soignants. La réflexion sur la fonction textile doit prendre en compte tous ces enjeux pour déterminer les organisations les plus adaptées. L'épidémie de Covid-19 et la gestion de la crise nous ont montré que l'organisation de la fonction textile avait une importance stratégique particulière, quel que soit le modèle retenu. Le nettoyage et la désinfection des textiles réutilisables sont des activités indispensables pour limiter les risques infectieux. Ils nécessitent un haut niveau de qualité et une grande réactivité. Nous devrons très prochainement analyser les différents modèles existants et en faire une analyse très précise pour assurer ce haut niveau de qualité attendu. Ces questions ont également leur place dans le Ségur de la santé, que ce soit dans les travaux nationaux ou dans les contributions qui parviennent des régions. Les activités logistiques sont partie intégrante d'une bonne organisation des soins : je souhaite que nous les intégrions dans nos propositions pour donner aux établissements tous les outils

En effet, très peu d'enfants en situation de handicap de moins de 3 ans sont accueillis par des assistantes maternelles : ils sont le plus souvent gardés exclusivement par leurs parents. Depuis le 1 novembre 2019, le complément de libre choix du mode de garde a été revalorisé de 30 pour les familles bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), afin de favoriser la garde des tout-petits, reconnaître le surcoût que peut représenter cette garde et, ainsi, assurer un meilleur revenu aux assistantes maternelles. Cependant, l'impact de cette mesure est limité sur 265 000 allocataires de l'AEEH, seuls 33 000 en bénéficient au titre d'un enfant de moins de 6 ans et 4 700 familles bénéficient de l'allocation pour un enfant et du CMG pour un autre de leurs enfants.

Le Haut Conseil proposait d'allouer une prime aux assistantes maternelles qui se formeraient pour accueillir un enfant en situation de handicap ou qui en garderaient déjà un. Quelles suites comptez-vous réserver à cette proposition de nature à favoriser la garde des enfants en situation de handicap par les assistantes maternelles ?

je vous remercie pour votre question, qui porte sur un sujet que je suis avec attention au ministère. La proposition du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge d'instaurer une prime pour les assistants maternels l'objet d'une expertise, mais, au-delà de cette mesure, beaucoup a déjà été fait pour rendre les modes d'accueil du jeune enfant plus inclusifs. En 2019, nous avons donné la priorité à la mise en place du bonus pour les établissements accueillant les enfants en situation de handicap, négocié dans le cadre de la COG entre l'État et la CNAF.

pour répondre aux besoins des parents d'enfants en situation de handicap, particulièrement éprouvés durant les mois de confinement. Par ailleurs, les travaux de simplification de la réglementation des modes d'accueil du jeune enfant, qui ont fait l'objet d'une large concertation, ont permis d'intégrer au projet le principe d'un renforcement de l'obligation des établissements à mettre en oeuvre le principe d'inclusion, ainsi que l'explicitation d'exigences dans la conception des bâtiments, telle que l'obligation de disposer d'un espace adapté à la réalisation de soins et d'un espace suffisant pour ranger le matériel nécessaire. Le projet d'instaurer dans chaque établissement un référent santé et inclusion, chargé d'accompagner les équipes et de renforcer les partenariats extérieurs, est conçu pour lever en partie ces freins. Il est également proposé d'expérimenter la mise en place de tels référents santé et inclusion au sein des relais d'assistants maternels de façon, là aussi, à accompagner les parents et les assistants maternels à l'accueil de ces enfants handicapés, toujours dans un souci d'inclusion. Enfin, le plan de formation des professionnels de la petite enfance retient l'accueil de la diversité comme un de ses six thèmes prioritaires. Sa mise en oeuvre auprès des 600 000 professionnels, dont les assistants maternels font partie, permettra d'améliorer l'accueil des enfants

Ces structures encadrées et contrôlées par le ministère des solidarités et de la santé répondent aux exigences réglementaires des politiques publiques de la petite enfance. À ce titre, elles bénéficient des financements des caisses d'allocations familiales, de même que les parents qui y placent leurs enfants. Elles accueillent environ 10 000 enfants, avec une forte concentration en Alsace, en Bretagne, à Paris et à La Réunion. Voilà un an, les jardins d'enfants ont été au centre des débats dans cet hémicycle. Le projet de loi pour une école de la confiance prévoyait leur suppression. Les échanges à l'Assemblée nationale et au Sénat ont permis d'élaborer un compromis leur octroyant un délai de cinq ans pour se transformer en écoles maternelles privées sous contrat ou hors contrat, ou se recentrer sur les enfants de moins de 3 ans. Lors de nos débats, Jean-Michel Blanquer déclarait : « L'État, au travers des plans de formation dédiés pour les personnels, pourra accompagner certaines structures qui le souhaiteraient vers leur transformation en école maternelle publique. » garder toutes les caractéristiques positives ». Or, près d'un an après l'adoption de la loi, les jardins d'enfants nous alertent sur le manque d'information et d'accompagnement.

Ces établissements sont, dans leur grande majorité et de manière significative, financés par les caisses d'allocations familiales, au même titre que les autres établissements d'accueil du jeune enfant. En abaissant l'âge d'instruction obligatoire à 3 ans, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance impose une évolution du fonctionnement de ces établissements, qui accueillent aujourd'hui des enfants de 2 à 6 ans. Les jardins d'enfants disposent néanmoins d'un délai de cinq ans pour s'adapter à ce nouveau cadre. L'intérêt pédagogique de ces structures est reconnu. Il nous faut donc préparer leur évolution au sein du nouveau cadre posé par la loi pour une école de la confiance. Par courrier du 3 janvier 2020, j'avais mandaté, avec Agnès Buzyn et Jean-Michel Blanquer, une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la jeunesse. Le 16 avril 2020, cette mission a rendu un premier rapport intermédiaire, qui a permis de conforter la connaissance de ces structures diverses et de faire état des différentes modalités de leur contrôle. La mission conjointe a également ouvert, le 3 mars 2020, une enquête auprès des responsables des jardins d'enfants, afin de recueillir des renseignements plus fins sur leur activité. Cette enquête viendra enrichir le rapport final de la mission, qui éclairera cette année les ministres, comme les établissements, sur les différents scénarios d'évolution possible de ces structures à l'horizon de 2024. La parole